Bonjour, chers collègues, bonjour monsieur le Ministre, la séance est ouverte, le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué, y a-t-il des observations. Je n'en vois point le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage j'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 1528 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 11 l'amendement 1528 Madame Espagnac. Oui, madame la présidente, merci Monsieur le Ministre, cet amendement, donc nous reprenons la discussion cet amendement vise à modifier les avantages fiscaux pour les entreprises de location de meublés touristiques, l'article 50 zéro du code général des impôts, porte un abattement forfaitaire de 71 pour ou 50 % sur les revenus de location de meublés de tourisme au titre du régime des micro-entreprises dans le cas où ces entreprises auraient un chiffre d'affaires inférieur 176200 176200 euros ou bien, soit 112600 euros, il propose de pardon, cet amendement d'exclure de ce régime fiscal les entreprises dont le commerce principal et la location de meublés de tourisme classé et ayant un chiffre d'affaires subir à 20000 euros, il propose également de créer une nouvelle catégorie pour les entreprises de location de meublés de tourisme non classés afin que seules celles il y a un chiffre d'affaires inférieur à 20000 euros contre 72600 aujourd'hui puisse baisser bénéficiant d'un abattement de 50 % l'esprit de cet amendement vise à ne pas encourager les locations de tourisme au détriment des locations longue à l'annexe qui est aujourd'hui un problème dans les Pyrénées Atlantiques, notamment au Pays basque, suffisamment donc pardon subissant un grave crise du logement, cette nouvelle disposition ne concerne pas les gîtes ruraux qui participent au développement local du territoire. Vous avez présenté les les deux chers collègues. Bien sûr, excusez-moi, madame la présidente, le second amendement donc vise à exclure les entreprises dont le commerce principal de la location meublée toujours pareil en zone tendue, les avantages qui prévu dans l'article 50 y'pardon, il vise aussi à ne à ne permettre un abattement que de 50 % pour les autres entreprises de meublés de tourisme à condition qu'ils aient un chiffre d'affaires inférieur à 72600 euros merci. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Monsieur le Ministre. Je mets donc aux voix c'est. Cher collègue Monsieur Lemoine pour explication de vote. Merci beaucoup, madame la présidente, effectivement, nous avons eu le le débat hier voilà par le le le du placement des amendements, nous l'avons à nouveau aujourd'hui et, pour être précis, hier justement Max Brisson portait aussi un amendement dans dans le même esprit, le gouvernement et et la Commission, on dit qu'il était ouvert à ce qu'un travail puisse avoir lieu sur cette base là et donc il me semble que les amendements que porte Frédérique Espagnac vont également dans le sens, hein, qui était, qui a été adopté hier et peuvent contribuer aussi au travail qui va être conduit dans les dans les prochains jours les prochaines semaines, puisque vous le savez, il y a une instance qui a été mis en place avec la secrétaire d'État à la ruralité avec le ministre du logement pour trouver des solutions justement et faire en sorte que, effectivement, la crise du logement qui touche certains territoires touristiques puisse encore une fois trouver un certain nombre de solutions, donc je trouve que nous pourrions également adopter ces amendements ça contribuera à ce travail qui va être conduit dans les prochains jours, sur la base d'autres amendements dans la même esprit qui ont été adoptées hier.

avec ce que nous avons voté avec l'avis de sagesse du gouvernement, il me semble en effet que l'amendement de Frédéric Espagnac complète celui que nous avons voté donc par cohérence au bras cas je le voterai puisqu'il va, il a le même objectif et il ouvre un chantier que Monsieur Attal a souligné et la navette nous permettrait, je crois, d'arriver à une solution, il s'agit bien aujourd'hui d'aller vers une fiscalité plus harmonisée, la situation actuelle est insupportable, il est plus avantageux aujourd'hui fiscalement de louer à l'année, il est plus avantageux aujourd'hui de soustraire au au locatif durable, les logements pour les mettre en location saisonnière, il me semble de bonne cohérence entre nous de suivre l'amendement de notre collègue. avec ces deux amendements avec 2 avis défavorable au vote. Qui vote pour. Qui vote contre. Alors on va refaire un qui va alors je mets le premier amendement parce qu'en fait c'est une discussion commune, ils sont pas identiques, je mets le premier amendement au vote le 1528 avec 2 avis défavorables qui vote pour.

Qui vote contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés. Le 1123 Monsieur Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, les obligations légales de débroussaillement autour des habitations 50 mètres en principe proche de la forêt constitue une mesure essentielle de prévention contre les incendies, permettant d'en diminuer l'intensité d'en limiter la propagation et de renforcer la défaite, l'habilité des habitations et aussi de protéger la forêt contre un accident domestique, elles sont malheureusement trop peu appliquée avec un taux de réalisation souvent inférieur à 30 pour inciter la réalisation des ALD le présent amendement prévoit l'instauration d'un crédit d'impôt pour dans le bénéficiaire serait subordonnée au respect des obligations envers la réalisation de débroussaillement par un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, et dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal, cet amendement constitue la traduction de la recommandation numéro 20 du rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie adoptée en août 2022, par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat, ce rapport montre que la protection de la forêt et les moyens de lutte contre les incendies ont le même intérêt pour éviter les feux de grande ampleur mais n'ont pas le même poids financier la notion de la valeur du sauver montrent que le ratio peut-être sur les territoires de un à vingt, d'où l'impact d'investir dans la protection de la forêt qui s'appuie sur 3 principes : principes principe à la main, la multiplication des pies DAF, il y a des pistes DFCI la politique de sylviculture pour enlever de la biomasse, de façon à ce que la forêt soit plus facilement défendable et surtout la généralisation des eaux il n'y a pas de recette miracle, mais la somme de nombreuses actions qui permettra d'être au rendez-vous du changement climatique et de ses conséquences. on va avoir plusieurs occasions de parler quand on regarde le l'objet de l'amendement dont je partage la préoccupation je vais demander donc l'avis du gouvernement, parce que j'ai, il y a je pense plusieurs sujets, il y a le débroussaillement proche du domicile il y a le débroussaillement forestier le montant qui est sollicité de crédit d'impôt est assez sensiblement inférieur, par exemple,

la réalité des situations, les orientations du gouvernement et les choix qu'favorise pour répondre à cette à ses obligations légales de débroussaillement dont on perçoit de plus en plus elles ne sont pas faciles, il n'est pas facile d'y répondre pour les particuliers, pas toujours facile d'y répondre, notamment lorsque, il y a des parties de forêt entre des habitations, donc avec des faibles densités d'habitat, mais également des risques importants qui sont liées aussi à la propagation de des incendies et pour terminer, il y a propagation des incendies et puis il y a respect de la biodiversité protection parfois des maquis des des justement de parcelles en broussaille et donc quelle possibilité vous prévoyez d'offrir aux particuliers pour qu'qui qu'il puisse répondre à ses obligations. Merci, Monsieur le Ministre pour explications sur ses préoccupations. Effectivement, merci madame la présidente, bonjour à toutes et à tous, on a évidemment une préoccupation partagée de lutter contre les feux de forêt, y compris en matière de prévention, ça concerne l'état, ça concerne les collectivités locales, ça concerne les particuliers qui ont aussi un certain nombre d'obligations et on parle ici du débroussaillage, vous le savez, on a pris un certain nombre de mesures dans le cadre de ce PLF c'est pas immédiatement liés à la prévention contre les feux de forêt, mais ça y participe, évidemment, notamment l'extension et le renforcement du défi forêt, il a par ailleurs des mesures très fortes qui ont été annoncées par le président de la République, il y a quelques jours un plan à 250 millions d'euros pour améliorer notre lutte contre les feux de forêt, il a 150 millions d'euros en 2023 sur les dix le renforcement de notre flotte de Canadair, là on a évidemment pas dans la prévention, mais dans le renforcement de nos moyens pour lutter contre les, il y a des situations très spécifiques que vous évoquez sur ce sujet-là, moi je pense qu'il faut qu'il y a un travail, je suis prêt, d'ailleurs amené avec lui, avec mon collègue Marc Fesneau, parce que ça dépend du ministère de l'agriculture en en l'espèce, pourquoi est-ce que je suis défavorable à la création de ce crédit d'impôt parce que je ne suis pas certain que ça soit l'outil le plus efficace et, par ailleurs, un crédit d'impôt normalement a une visée incitative pour inciter à réaliser quelque chose ou à réaliser une action en l'occurrence, là on parle d'obligation légale de créer un crédit d'impôt pour ce qui relève d'une obligation légale ne ne semble pas vraiment et dans la philosophie du crédit d'impôt qui, normalement, une visée incitative, précisément pour des, des, des, des, des, des actes ou des décisions qui ne sont pas obligatoires, donc sur le dispositif en tant que telle, avis défavorable en revanche sur la nécessité d'aller plus loin, comme on l'a fait avec le renforcement des moyens des collectivités territoriales, des moyens de l'État, d'aller plus loin avec peut-être de nouvelles initiatives en direction des particuliers, là je vous rejoins totalement et je suis prêt à travailler avec mon collègue Marc Fesneau.

on parle d'eau LD les Zolder c'est 50 mètres autour de la maison, donc il s'agit pas d'aller en forêt, il s'agit pas d'écarter et de de promouvoir des travaux forestiers, on parle de protection des biens et de protection des des personnes surtout j'étais corapporteur avec mon collègue Jean Bassim mais également Pascal Martin et Anne-Catherine Loisier sur la mission pour limiter l'extension des feux, il ne serait pas utile et même contre-productive d'annoncer des dépenses de millions de milliards des bateaux, des bateaux, des véhicules pour intervenir sur les grands feux si on n'applique pas la base même de la lutte contre les incendies, la protection des biens et des personnes, quand on a commencé notre mission, on a fait un déplacement dans le Var pour analyser les conséquences du grand feu de Gonfaron et quand on voit des vues aériennes du feu de Gonfaron c'était plus de 20000 hectares, on se rend compte que les seuls petits points verts qui subsistent au milieu de tout ce qui a été brûlé, c'est là où les Zolder ont été faites à la perfection, 50 mètres autour des habitats, le seul endroit où il y a eu un décès, c'est une maison autour desquels il n'y avait aucune nouvelle des qui avait été fait il est impossible, si je reprends les paroles du contrôleur général Grégory Allione de mettre un camion de pompiers derrière chaque maison dans un habitat diffus dans ces secteurs là d'un j'en veux avec les la présence d'un camion de pompier et empêche de mobiliser les pompiers sur une habitation, elle leur permet d'aller lutter contres les feux en forêt cet cet engagement d'LD est primordial, je vous demande vraiment cher collègue de nous suivre sur cet amendement, il engage pas énormément d'argent, d'autant plus que si on prend le coût du sauver toujours les paroles de Grégory Allione 200 millions engagés dans la lutte contre les incendies ces dernières années, 5 dernières années dans le le Sud et Sud-Est ont engendré d'après les études, plus de 5 milliards de sauver de bâtiments de d'entreprise et de biodiversité, ça sera plutôt une économique, une dépense d'argent merci. Oui, mes chers collègues, moi je, j'entends les arguments mais je, je, je trouve qu'il y a un lien qui est fait, si vous voulez entre un sujet qui est réel, une présentation du dossier impeccable, chers collègues, qui pose pas de problème intellectuel et la réponse qui est apportée d'abord quand il a une obligation légale, comme le disait le ministre quand il y a une obligation légale, venir soutenir les populations pour remplir une obligation légale de cette nature qui est quand même pas non plus quelque chose d'extraordinaire que d'entretenir cinquante autour de son habitation, je, je, je pense même que pour les maisons qui sont dans dans des zones de forêts même des clauses d'assurance doivent obliger à le faire et qu'il y a pas de remboursement, si vous le faites pas, enfin vous moi je pense que des gens qui n'entretiennent pas leur tour de maison alors qu'ils ont une obligation de le faire d'une part et d'autre part qu'ils ont un intérêt personnel à le faire, je ne vois pas pourquoi l'État viendrait soutenir avec l'argent public et d'ailleurs, même si le mettez-moi si les gens veulent pas le faire, c'est pas parce qu'il y a une aide, une aide financière qu'ils le font plus, enfin voilà, donc moi je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt le la question a beaucoup d'intérêts, excusez-moi, hein, chers collègues, mais la réponse n'est pas adapté. Monsieur le rapporteur, nous avons donc un avis défavorable du gouvernement votre avis. Ce sera un avis de sagesse pour faire avancer le dossier. Monsieur le ministre. Ah d'accord j'émets donc on voit cet amendement avec cannabis sagesse de la commission défavorable du gouvernement qui vote pour.

eu égard à la situation économique du pays, la mutualisation de personnel à but non lucratif particulièrement via le dispositif groupement d'employeurs régis par le code du travail apparaît désormais indispensable les groupements d'employeurs, occupe une place à part dans les dispositifs de prêt de main-d'oeuvre en favorisant des emplois durables, ils ont trouvé au fur et à mesure des années, et particulièrement à l'occasion de la crise de la Covid 19 qu'il pourrait s'adapter aux différentes situations économiques et sociales, qu'il s'agisse de périodes de crise ou de croissance, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit donc dans son article 45 la modification de l'article 261 B du code général des impôts, il s'agit là d'une véritable occasion de confirmer le soutien au Sénat du Sénat auprès de main-d'oeuvre, comme le prévoit le plan de relance, particulièrement au groupement d'employeurs qui organise et sécurise ce prêt en effet la question du régime TVA fait partie des au vu des évolutions indispensables pour des le voeu Lopé les groupements d'employeurs lorsqu'un groupement interviennent à la fois auprès d'associations ou de structures non soumises à la TVA et auprès d'adhérents soumis à TVA il est soumis à la TVA sur l'intégralité des mises à disposition, la facturation de TVA, c'est à des structures qui ne peuvent la récupérer constitue un frein considérable à l'adhésion de structures principalement des associations et des collectivités territoriales, cela empêche ainsi de compléter le temps de travail, de nombreux salariés et oblige la crème à la création de ce groupe, hein, bande d'employeur à destination exclusive d'adhérents non soumis à la TVA, nous demandons donc la possibilité de ne soumettre à TVA que les mises à disposition auprès d'entreprises soumises elles-mêmes à TVA, cet amendement est un amendement de notre collègue Nathalie Delattre. Merci de l'avoir brillamment défendu, chers collègues, monsieur le rapporteur. je vais avoir le plaisir de vous dire de vous proposer le retrait mais pour une bonne raison, c'est qu'il est satisfait par l'amendement 644 que nous avons adopté hier et qui était présenté par le sénateur Pell va.

ce qu'il en sera dans la suite de la navette et donc je vais être très clair sur le fait que non seulement il est manifestement satisfait par cet amendement, mais cet amendement est aussi satisfait par la doctrine fiscale puisque la question qui est posée avec cet amendement, c'est est-ce que dans un groupement de moyens, si un des membres est assujetti à la TVA est-ce que ça fait tomber le groupement de moyens est ce que elle peut ne pas être prélevées dans des services entre membres du groupement de moyens quand bien même il y en a un qui assujettis à la TVA, la réponse est oui c'est précisé dans la doctrine fiscale l'assujettissement à la TVA d'un des membres ne fait pas tomber le groupement de moyens et donc je tenais à être clair, quel que soit le sort réservé dans la navette à l'amendement 600 cent quarante-quatre c'est satisfait par la doctrine fiscale. Si vous retirez merci. L'amendement 1333 monsieur le Président, Ruquier. Merci madame la présidente, monsieur oui, mes chers collègues, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté l'article 5 l'alignement de l'exonération de la taxe d'habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, à l'image de celle dont bénéficient déjà les structures du secteur public assurera les mêmes émissions avec les mêmes modalités de si aisément de leurs charges dans la taxe d'habitation à l'état algérien utilise cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches, s'agissant des obligations auxquelles ils peuvent être soumis le concours, notamment pour le coup de l'hébergement au regard des règles relatives à l'aide sociale de l'État ou des conseils départementaux à l'écoute, cette demande légitime le gouvernement à l'Assemblée nationale en cause ça en seconde lecture,

d'intérêt général que le Sénat avait décidé d'exonérer dans leur globalité, à l'image des structures publiques, telle est l'objet, c'est au mois de novembre Nathalie Delattre qui étend le périmètre concerné et apporte les gages nécessaires à cette extension. Monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Donc pour cet amendement qui, qui a le la vertu de proposer une exonération obligatoire non compensées, si ce n'est pas compensé ça veut dire que c'est une perte de recettes pour les collectivités territoriales, vous savez qu'on est plutôt attaché à la au maintien de nos recettes, donc je, c'est un avis défavorable.

les installations de stockage de déchets ISD sont conçues pour traiter des déchets ménagers ou d'activité économique dans des casiers aménagé à cet effet, et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l'environnement. Une ISD. est ainsi constitué de plusieurs casiers exploiter l'an après l'autre, indépendants des uns des autres est conçue de façon à permettre la des effluents générés par cette activité. Dans la rédaction actuelle, l'article 499 00 ah prévoit que la modification de l'évaluation des valeurs locatives doit avoir lieu après la couverture finale du dernier casier or USD est composé de plusieurs casiers qui sont exploités durant une période de un à 2 ans, ainsi la couverture du délai casier peut avoir lieu plusieurs années voire plusieurs décennies après le début d'exploitation de l'ensemble du site dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISD peuvent être équipés de panneaux photovoltaïques sur ces casiers fermé qui présente des caractéristiques techniques optimales et limite ainsi l'artificialisation de surface naturelle pour le développement du projet solaire une première estimation réalisée par des acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 à l'horizon 2040 le présent amendement a donc pour but de permettre une modification de l'évaluation financière casier par casier et non pas à l'échelle de l'ensemble du site comme ce ce aujourd'hui, je vous remercie. Mais comment dirais-je, mettent sous le projecteur des situations dans lesquelles on va se trouver avec des objectifs en temporalité. De, comment dirais-je, d'investissement et de dispositifs qui porte l'un comme l'autre des préoccupations environnementales site pardon hier de stockage de déchets aujourd'hui ou demain, installation de panneaux photovoltaïques, l'objet de l'amendement et d'essayer de rendre plus favorable. Pour certains, en tous les cas, le dispositif, c'est l'objet de l'amendement, mais je note. Que dans le même temps, la disposition, elle peut avoir des difficultés techniques de mise en oeuvre et qu'elle conduit aussi à avoir un impact à la baisse sur les recettes des collectivités territoriales, donc pour faire clair, la problématique s'inscrire dans la temporalité de la transition écologique et énergétique et puis répondre aux enjeux et comme l'a dit le sénateur chaises en plus de d'être quasiment à la fermeture et au traitement de du retrait des casiers de stockage au fur et à mesure du temps pour avoir la meilleure adéquation entre ce qui est perçu, et qui est évidemment plus onéreux quand on est en site de stockage et ce qui est perçu au bénéfice des collectivités territoriales, s'agissant de ses impôts, quand ce sont des installations photovoltaïques, Monsieur le Ministre, nous avons donc besoin de votre avis. Merci, alors Monsieur le Ministre votre avis. à limiter au stockage de déchets non dangereux ce dispositif compte tenu des expertises, des installations il était manifeste, il semblait manifeste à l'époque où cette décision a été prise, que le besoin était limité à ces installations là le dispositif actuel nous semble être un équilibre en ce qu'il permet de ne pas avoir une taxe foncière excessives pour ses activités tout en préservant les ressources des collectivités locales, donc nous on souhaiterait en rester à cet équilibre, j'ajoute que dans l'amendement qui est proposé, le dispositif juridiquement ne nous semble pas tourner totalement puisque, en terme de notification au titre des ICPE, il représente un problème opérationnel de procédure, comme ça a été sous-entendu par le rapporteur général pour ces raisons avis défavorable, monsieur le rapporteur. Votre avis défavorable très bien je mets donc cet amendement envoient avec 2 avis défavorables qui vote pour.

mais qui dit j'dit vas-y un petit peu les installations de stockage de déchets sont conçus pour stocker des déchets ménagers ou d'activité économique dans des casiers aménagé pour sa TV et j'ai des pourraient être équipé de panneaux photovoltaïques sur les casiers, on pense exploitation,

qui ont du prix de revient ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou propriété comprenant des équipements souterrains indissociable des casiers, des installations de stockage des déchets à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'achèvement de la couverture finale du dernier casier de l'installation de stockage a été notifié par l'exploitant à l'inspection des installations classées, oui, c'est très clair, il n'a entendu ce n'est que que lors de la session de toute activité là officiellement qu'il est possible de constater le changement d'affectation et dans le passage d'une activité industrielle à l'activité professionnelle, le président propose de permettre aux projets photovoltaïques de bénéficier du changement d'affectation prévue dès la libération des terrains d'accueil, tu as le droit, Alain Madelin, qui a été travaillé avec le syndicat des énergies renouvelables. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. J'avais prévu un avis du gouvernement, le gouvernement vient de répondre assez clairement à la à l'amendement précédent du sénateur, chaises, c'est donc un avis défavorable. Monsieur le Ministre, même avis. Retiré. 5 amendements en discussion commune Monsieur Breuiller le 605. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, notre amendement vise à établir la taxe de séjour non plus selon un montant fixe comme c'est actuellement le cas, mais en pourcentage du prix de la nuitée actuellement la taxe de séjour avec un montant fixe a des conséquences négatives sur les établissements hôteliers hôtel de plein air, proposant des prix bas, dans la mesure où cette taxe représente une part de dépenses plus importantes pour les clients que pour les établissements hôteliers proposant des prix plus élevés, nous proposons donc de modifier l'échelle de tarif fixe par catégories d'hébergement en permettant aux collectivités et c'est encore une volonté de leur donner plus d'autonomie, de définir des tarifs proportionnel au prix de l'annuité dans une fourchette de 1 à 7 pour 100 du montant facturé sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme. Merci Monsieur Féraud. Lech, vous pouvez présenter les deux oui s'il vous plaît, tout à fait, nom mon nom de repli. Concerne également la la taxe de séjour pour vous montrer les les enjeux que cela représente, c'est à peu près 500 millions d'euros en année normale, c'est-à-dire hors Covid et ça représente c'est est perçu sur à peu près 3000 collectivités bien évidemment

proportionnalité de la manière dont on vient d'évoquer le le collègue précédemment et s'agissant du et pour pour la taxe pardon pour la taxe réel effectivement de la proportionnelle Izé en appliquant un taux sur sur les tarifs d'hébergement et s'agissant de la taxe forfaitaire, la proposition qui est faite simplement c'est de relever les fourchettes de tarification en les doublant l'amendement de retrait reste dans l'esprit de la taxe aujourd'hui du régime telle qu'il est appliqué, avec simplement une revalorisation des de, de, de la fourchette de taux dans lesquelles les collectivités doivent fixer les tarifs applicables sur leur territoire. Merci, monsieur le sénateur, joli, l'amendement 193 monsieur le sénateur Brisson. Merci madame la présidente au monde amendement et ce qui précède et ont été propose que le tarif proportionné applicable aux hébergements hors classement, c'est-à-dire entre autres aux meublés de tourisme non classés soit aligné sur le taux le plus haut voter dans la grille tarifaire, il s'agit d'harmoniser les conditions de la concurrence pour l'hôtellerie et les hébergeurs professionnels. Merci madame la présidente, aujourd'hui le tarif applicable aux croisiéristes en matière de taxe de séjour ne tient absolument pas compte de la prestation hôtelière des navires d'une qualité bien supérieure au terrain de camping et terrains de caravanes classé en 1 et 2 étoiles auxquels ils sont assimilés jusqu'à présent, il ne tient surtout pas compte de leur impact environnemental, souvent à la charge des collectivités, de nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution importants générée par les paquebots et les navires qui utilise à fioul lourd dont la teneur en soufre et 3500 fois supérieurs aux normes tolérées pour les sciences terrestres cet amendement permettrait ainsi aux collectivités d'augmenter la taxe de séjour qui s'applique aux navires de croisière les plus polluants grâce à une majoration jusqu'au tarif plafond de 10 euros les navires utilisant l'hydrogène ou toute autre proposition décarbonés pour être évidemment faire l'objet d'un traitement particulier c'était initiative ne vise pas à pénaliser le secteur du tourisme déjà fortement meurtri par la crise sanitaire et économique aussi, dans un souci de neutralité fiscale, nous proposons d'abaisser de 10 % le tarif plafond de la taxe de séjour qui s'applique aux hôtels de tourisme 1 2 et 3 étoiles ainsi qu'au terrain de camping et aux emplacements de camping car. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis sur tous ces amendements s'il vous plaît. Voilà donc des amendements qui touche tous le même sujet où il y a, je dirais une certaine forme de créativité, mais pas d'accord que sinon ils auraient été tous identiques, donc le l'arbitrage que je vous propose et de un avis de sagesse pour le l'amendement 193 actif bis déposé par le sénateur Brisson, une demande de retrait pour les 4 autres amendements au profit justement de cet amendement 193. Merci, Monsieur le Ministre votre avis. Merci, c'est un sujet qui revient régulièrement dans des débats budgétaires, et je pense qu'il faut être assez clair sur le sens du débat et le fond du débat, c'est une mesure qui est parfois, je ne dis pas que c'est le cas ici, hein, mais souvent dans le débat public quand elle est avancée, qui est parfois avancé comme une forme de mesures symboles Taxer les palaces, je considère pas que la fiscalité soit un outil de symboles, c'est un outil de redistribution je crois pas que ça soit un un outil avec lequel il faut faire du symbole, sinon on trouvera toujours beaucoup de symboles et à la fin, ça finira par frapper et toucher beaucoup de monde, ou alors dans certains cas c'est mis en avant comme une mesure qui permettrait d'équilibrer le budget de certaines collectivités très endettées et là non plus, ça ne peut pas être le cas, il veut pas faire croire qu'avec une augmentation du plafond sur la taxe sur les palaces dans une grande collectivité qui bénéficieraient de beaucoup de palace, ça change la donne, quand on compare le montant du besoin de financement des déficits et de la DS et la dette avec le montant que rapporterait une taxe sur la dizaine ou un peu plus de palace dans cette collectivité donc moi c'est pour ça que je suis assez réservé sur ce sujet-là, il y a aussi une question de symbole envoyé dans la concurrence entre guillemets entre les pays touristiques européen et sur le niveau de taxation qu'ils appliquent à leurs hôtels, encore que pour quelqu'un qui peut se payer une grande fuite dans un grand palace, on peut toujours se dire évidemment que c'est pas le niveau de la taxe de séjour ou du plafond qui va particulièrement jouer sur son envie de venir à Paris, à Paris ou pas, par ailleurs pour un certain nombre d'amendements qui ont été présentés, il y aurait un effet de bord puisque ça ne relèverait pas le plafond uniquement sur les palaces, mais sur l'intégralité des hôtels non classés et donc y compris sur des hôtels qui n'ont rien à voir avec des palaces et le risque oui, mais le risque c'est qu'à la fin ça aussi un effet négatif défavorables en matière touristique pour le coup, si ça touche des hôtels ou des nuitées qui n'ont rien à voir avec des grandes fuites dans des grands palaces, mais qui concerne des hôtels plus modestes en tout en tout cas pour des touristes donc pour ces raisons-là avis défavorable. Merci Monsieur Féraud pour explications de vote. Merci madame la présidente, il y a plusieurs amendements qui vont dans le même sens, même si leur mécanisme sont légèrement différents je remercie monsieur Brisson d'avoir déposé cet amendement, ce que j'ai bien entendu le ministre qui pense beaucoup à Paris répondre en pensant à Paris mais il ne faut pas que ce soit une obsession et il faut que ce soit aussi pour l'ensemble de nos collègues, une alerte, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le débat que nous avons eu hier sur les résidences secondaires les meublés de tourisme moi comme sénateur de Paris avec d'autres sénateurs de Paris et d'Île-de-France, cela fait longtemps que nous alertons sur les difficultés de se loger, pour les habitants d'un territoire et parfois on nous regarder avec un peu d'indifférence mais aujourd'hui ces questions ces enjeux d'accès au logement se sont développées sur beaucoup de territoire français et nous n'avons pas les mécanismes pour l'empêcher le limiter et permettre à la fois aux collectivités d'avoir des ressources, c'est vrai, mais aussi aux personnes de se loger, il s'agit bien des 2 sujets toujours à la fois donc j'entends l'attractivité touristique, et cetera enfin rechercher sur Internet, le prix d'une chambre de palace à Paris, c'est plusieurs milliers d'euros la taxe de séjour aujourd'hui limité à cinq euros il y a des amendements qui propose la l'augmenter jusque vers huit dix euros, ça dépend des mécanismes bref ça ne crée aucun problème d'attractivité touristique en revanche, ce sont des ressources supplémentaires pour les collectivités, ce qui évitera d'augmenter d'autres impôts qui pèsent sur les habitants et puis c'est aussi par le mécanisme sur les meubles et Tourisme, une façon de préserver l'accès au logement des habitants des territoires, donc j'espère que, au moins l'un de ces amendements pourraient être adoptées aujourd'hui, ça n'est pas qu'un symbole, c'est aussi une mesure très concrète et le symbole, il est positif Monsieur le Ministre. Là que vous retirez les de votre vous voulez laisser au vote d'accord Monsieur Lemoine pour explication de vote. Merci madame la présidente, sur les, les, les amendements que vient de présenter, Rémi Féraud, un point d'attention puisque ce calcul en pourcentage il n'est pas que pour la catégorie Palace et dans le tableau, il est pour l'ensemble des catégories et la France, c'est une destination touristique, pas que pour le loisir, mais également une destination pour le tourisme d'affaires pour le tourisme d'affaires, prenons garde à ne pas pénaliser la destination France, pour le coup, parce que les acheteurs si je puis dire, les sociétés qui organise des séminaires, des salons, des foires et sont très attentives, pour le coup à la compétitivité et et donc on voit bien l'esprit qui préside aux amendements mais mais je voulais signaler ce point qui doit nous inciter à être très prudents dans, dans, dans, dans la façon dont on aborde le débat, je relève d'ailleurs que l'amendement justement de, de, de Max Brisson

je veux dire, parce que il ne faut pas qu'on qu'on croit que l'industrie de la croisière reste les 2 pieds dans le même sabot, il y a véritablement une détermination à aller vers un tourisme plus durable, d'ailleurs les ports s'équipe, c'est le cas à Marseille pour que les navires puissent se recharger de, de, de, de, en, en électrique éviter effectivement les pollutions et et je voulais le site à ce moment-là du débat parce que on entend toujours effectivement un certain nombre de reproches, mais ce sont des acteurs qui aussi cherche à se transformer et et et à aller de l'avant, voilà les éléments que je je voulais porter à la connaissance de notre assemblée, la présidente. Merci monsieur Brice, explications de vote. Merci madame la présidente, moi je voudrais dire à monsieur le ministre, qui n'est plus là, que je n'ai. Aucune hostilité ben attendu. Oh. Excusez-moi, donc je, je, je, rapidement, c'est-à-dire que j'ai une bien sûr aucune hostilité pour les hôtels de grande qualité des hôtels de luxe, ni même pour les palaces, puisque j'ai été élu pendant 23 ans d'une ville qui possède un pas un palace qui est l'hôtel du Palais, dont une partie des travaux de rénovation avait été d'ailleurs été été inaugurée par Jean-Baptiste Lemoyne, lorsqu'il était secrétaire d'État au Tourisme en fait ce que le sens de mon amendement c'est d'harmoniser. La fiscalité qui porte sur les meublés de tourisme non classés avec la fiscalité qui porte sur l'hôtellerie, aujourd'hui il faut laisser la possibilité aux communes de pouvoir utiliser toute la palette de taxation de l'hôtellerie pour éventuellement aussi monter la taxe de séjour de certaines de tourisme au niveau de cette de celle des palaces et il s'agit d'une ou quelque quelque chose qui est attendu par là pour pas la profession hôtelière qui est aujourd'hui dans une situation de distorsion de concurrence, y compris aujourd'hui celle de de l'hôtellerie de qualité par rapport à certains meublés de tourisme, donc ce que l'on demande simplement à travers cet amendement c'est une harmonisation et je vous invite mes collègues à la voter après l'avis de sagesse que du rapporteur dans et je remercie.

Je voudrais saluer l'arrivée de de madame la Ministre bonjour et donner la parole pour explications de vote au président la font. Oui, juste pour dire que je le maintiendrai mon amendement parce qu'il est né d'une nature un peu différente de celle de mes prédécesseurs et et singulièrement de de celle du sénateur Brisson je voterai celui du sénateur Brisson moi ils portent plus exclusivement sur la question des des navires polluant et je parlais bien des navires polluants, vous avez raison, Monsieur le Sénateur Lemoine qui a, il y a, il y a des navires qui font des efforts de reconversion, mais il y en a encore qui utilisent du fioul et et on sait tous, l'impact environnemental, que ce type de de bateau peut peut avoir donc c'était cela qui étaient concernés dans mon et c'est donc un amendement d'une nature différente certes, ça porte sur la taxe de séjour mais il il est un homme à mon point de vue non pas complémentaire mais de nature différente à ceux de mes prédécesseurs. Merci Monsieur Bruillet vous retire votre amendement comme demandé ou pas très bien je mets donc aux voix l'amendement 605 avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre. Abstention : il n'est pas adopté, je mais aux voix l'amendement 555 avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre. Abstention : il n'est pas à adopter, j'estime que le 556 le même vote, je mets donc aux voix l'amendement de 193 avec donc un avis de sagesse, monsieur le rapporteur, et un avis défavorable du du gouvernement qui vote pour.

Toute émue du succès de votre amendement précédent allez-y monsieur le sénateur. Merci madame la présidente, Non, non je pense pas, nous étions plusieurs à raconter, donc il y a pas de souci, monsieur Brisson Alesi sur le 192. fiabilité, l'utilité et l'effectivité des États déclaratif de taxes de séjour transmis aux collectivités locales par les longueurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les plateformes de location meublée aussi les temps il encadre les périodes de référence utilisé pour les reversement de la taxe de séjour en effet si les textes fixe le calendrier de reversement de la taxe, il n'est en rien il ne coupe rien ne concerne les plages de référence, les collectivités reçoivent aujourd'hui des déclarations hétérogène, rendant plus difficile : Contrôle et exploitation statistique. Monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. C'est une une de c'est pardon c'est une demande de retrait parce qu'en fait il nous paraît qu'il y a des vraies difficultés de mise en oeuvre, notamment quand tu les réservations se font très en amont et ensuite pour le recouvrement parfois, ça devient compliqué lorsque il faut faire les reversements ultérieurement une demande de retrait. Merci, Madame la Ministre, pardon, excusez-moi, le temps est le changement. Bonjour, madame la présidente bonjour mesdames, messieurs les sénateurs. Gounod non monsieur le sénateur Brisson puisque et Gounod n'est ravi de vous retrouver, comme l'a dit le rapporteur à l'instant, on a sur votre proposition en réalité un un problème lié au au calendrier de reversement la loi et là, très clairement précisées les dates de reversement aux collectivités et il a été choisi de ne pas fixer la période concernée, pour justement laisser au collecteur le soin de s'organiser, l'essentiel étant que de reversement couvre 12 mois de collecte et toutes les plateformes, techniquement, n'ayons pas les mêmes moyens informatiques humain ça paraît difficile d'aligner le calendrier pour toutes et et par conséquent encadrer les périodes de collecte de la taxe de séjour complexifierait voir ne pourrait ne pas fonctionner en en matière de reversement de la taxe pour ces raisons, je vous demanderai de retirer l'amendement, le cas échéant, ce sera un avis défavorable je vous remercie. Monsieur Brisson pour explication de vote. Oui, madame la présidente, je vais retirer cet amendement mais je voudrais quand même signaler qu'il y a un problème parce qu'aujourd'hui les plateformes joue sur cette absence de référence du calendrier de déclarations et que cela n'est pas à l'Avantage des collectivités, il y a un véritable poubelle alors comme la commission et le gouvernement ont été plutôt favorable, avec l'ensemble des amendements que j'ai pu déposer depuis hier concernant le sujet des meublés de tourisme et que j'ai ressenti de la part de la Commission et du gouvernement une véritable écoute, je vais le retirer mais s'il reste un problème, cet amendement avait été d'ailleurs travailler avec la Commission des directeur des services financiers, des communes touristiques qui considère bien aujourd'hui qu'il y a une perte en ligne dans la collecte de la taxe de séjour et que cela mérite un vrai travail qui sera menée dans le cas de la commission dont parlait d'ailleurs Jean-Baptiste Lemoyne hier. Merci, cher collègue Madame Berthe et je vous engage à présenter vos deux amendements, si c'est possible. Merci oui, madame la présidente, c'est ce que je pensais faire effectivement madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, ces amendements visent donc tous les deux à permettre la vente d'huiles végétales usagées ou issus des graisses et autres résidus à l'exception de l'huile de palme comme carburant pour une utilisation précise-t-elle que l'aménagement et l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, grâce à cette inclusion ces biocarburants avancés comme le HVO 100 bénéficieront d'une baisse majeure de leur taxation le HVO sont, par exemple, permet de réduire de 80 % les émissions de CO2 selon l'Ademe et les professionnels du secteur, mesures une réduction de 60 % des émissions de particules fines par rapport au diésel, le régime fiscal actuel ne permet pas de prendre en compte cette solution majeure dans le combat contre les émissions de gaz à effet de serre alors qu'il s'agit ici d'une démarche très vertueuses, tant au niveau économique qu'au niveau écologique, notamment pour les activités de la montagne montagne qui doit pouvoir continuer à innover afin de répondre au mieux aux enjeux climatiques. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Oui, pardon, ce sera une demande de retrait sur ce type de carburant pour 95 % ils intègrent encore aujourd'hui de l'huile de palme. Donc il faut faire attention, alors on a toujours la question du levier fiscal et ce qu'il est décisif ou pas. Souvent non parfois oui, en tout état de cause, comment dirais-je, je pense qu'il nous faut avoir davantage d'éléments de connaissance et d'analyses pour apprécier la pertinence du dispositif dans votre amendement, vous visez des carburants qui aujourd'hui n'ont pas atteint leur seuil de maturité et d'ailleurs ils rejoignent un des cas que j'avais évoqué je crois hier ou dans la nuit précédente, ils sont aujourd'hui observé par des flottes captives enfin et sur le fondement d'une étude d'impact, je pense qu'il pourrait s'avérer qu'une telle mesure pourrait aller d'ailleurs au-delà si elle doit prospérer en fonction de, c'était une dévaluation du seul entretien des pistes ou des routes de montagne, mais en attendant, une demande de retrait. je le retire, mais effectivement je pense qu'il y a un un suivi à faire et une avancée à faire dans ce domaine. Vous les deux oui les deux pardon je voulais quand même dire un mot, Madame la Ministre, sont retirés. Je vous remercie, madame la présidente j'ai manqué de réactivité, je voulais juste j'avais levé un peu la main avant ces amendements à l'endroit du cent quatre-vingt-douze de monsieur Brisson, qui a été retiré, avant que vous ne Filliez juste vous dire que le sujet sur la taxe de séjour est un sujet qu'on est prêt à travailler avec les équipes de Gabriel Attal. à bon entendeur, n'hésitez pas à nous solliciter, je vous remercie. Merci madame la présidente, moi je voulais rebondir sur les les trois amendements, je crois que j'ai dit une à trois, je les ai lus de de Madame Berthet, qui ont le mérite d'exister et de rouvrir, Madame la Ministre, un débat qu'on a déjà eu au moment de la loi, pouvoir d'achat sur les huiles usagées et les constructeurs, les motoristes, les avionique se pose des questions, mais il commence à y travailler, et il y a pas de filière en France et il y a peut-être quelque chose à gratter là-dessus, même si c'est 5 10 % % à l'heure où on cherche tous les moyens d'énergie possible ce qu'a soulevé notre collègue Martine Berthet aujourd'hui c'est vraiment quelque chose à travailler, ce que je suis convaincu qu'il y a quelques niches potentiellement de ressources en énergie et en carburant, merci madame la présidente. Prime madame Berthe et le 776. Oui, donc il est toujours madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur général sur le même sujet, et celui-ci vise à inclure dans l'article 265 terre du code des douanes c'est et dans le Champ des carburants non roulant donc ces huiles végétales usagées ou issues de graisses, et cetera et comme vient de le dire, mon collègue, effectivement, nous devons donner un signal aux industriels afin de créer une filière française dans ce domaine et nous en avons vraiment besoin. Merci, monsieur le rapporteur. C'est vrai, mais votre amendement vise des dispositions du code des douanes qui sont aujourd'hui pour ce motif, je vous propose ou je demande le retrait.

Merci madame la présidente, madame la ministre, l'extension de la TASCOM aux entrepôts de commerce électronique est régulièrement proposés mais à ce jour la mesure n'a pas encore été retenus par le gouvernement, il faut pourtant contrer la concurrence déloyale dont souffrent le commerce de proximité, pourtant essentiels à la vie de nos communes et territoires face au commerce en ligne dans une situation d'urgence économique et social, cet amendement vise à rétablir un peu d'équité entre commerce de proximité et plateformes de E-commerce, les quelques mesures qui ont été prises pour tenter d'instaurer un meilleur équilibre entre la taxation du commerce physique et celle du commerce en ligne ne sont pas opérantes comme le monte la position toujours plus dominante des géants du E-commerce étrangers en France et la destruction de 85000 emplois en 10 ans dans le commerce physique cet amendement propose donc de soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, les acteurs du commerce électronique via la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés comme magasin de commerce de détail mais au départ desquels hé bien sont livrés directement ou indirectement, à travers des entrepôts de transit à destination des personnes physiques avec cet amendement, la TASCOM et du quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui exploite ces entrepôts dès lors que son chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 460000 euros. Merci, monsieur le rapporteur. Il me semble que l'amendement telle qu'il est rédigé aujourd'hui ne fonctionne pas vraiment pour ce votre proposition de la TASCOM aux entrepôts de stockage parmi les difficultés identifiées, il y a notamment le risque d'une double taxation puisque dès lors que les entrepôts peuvent aussi servir au stockage de bien finalement consommer dans un commerce assujettis à la TASCOM et pour les acteurs visés il y a en plus à risque, c'est que cette taxe devienne assez facilement contournable par le biais, par exemple d'une externalisation des dépôts partout où c'est possible, juste à l'extérieur de nos frontières, un avis défavorable. Merci madame la Ministre. Merci madame la présidente j'ai à coeur de de partager sur cet amendement 1082 un point qui me semble important en tant que ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. C'est un vrai sujet. Et par ailleurs, comme c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui sera traité dans les priorités. Du conseil national du commerce, qui sera mise en place, comme je l'ai annoncé il y a quelques semaines à la suite de la demande unanime et légitime des acteurs du commerce d'être présenté au sein d'un conseil national, il y aura des travaux sur l'équité fiscale qui viendront d'ailleurs compléter les travaux qui ont déjà été fait, vous le savez, sur la TASCOM relatives à l'équité entre les commerces physiques et les commerces digitaux, je vais vous dire que si, aujourd'hui, à cette heure, on n'a pas encore trouvé techniquement les voies et moyens pour ne pas taxer comme l'a dit le rapporteur par 2 fois les mêmes entités ne pas taxer, là ou les entrepôts des grandes surfaces ne sont pas d'accès certains acteurs français en gros la mesure elle est fondée, mais aujourd'hui on n'arrive pas encore à la faire avancer, je veux quand même vous dire à quel point j'en fais un sujet au coeur du conseil national du commerce et c'est une invitation monsieur le le sénateur à travailler ensemble sur ce sujet puisque, je le redis, la légitimité de la mesure me semble fondée, maintenant faut qu'on trouve les moyens pour que ce soit équitable et que ce ne soit pas une énième mesure fiscale facilement contournable, comme l'a rappelé le rapporteur, ce qui n'est pas encore le cas ce sera donc un avis défavorable, une demande de retrait, un avis défavorable, mais aussi une invitation et un rendez-vous dans les mois qui viennent à y travailler à nouveau ensemble pour qu'on trouve un atterrissage, je vous remercie. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues Madame Nice accueille avec beaucoup d'intérêt vos propos parce que ça fait de nombreuses années qu'ici même, nous revenons avec les mêmes amendements ou des amendements voisin sur la TASCOM sur la la taxation éventuelle des livraisons également avec des versions toutes différentes et à chaque fois, nous avons les mêmes arguments non dépourvue de pertinence d'ailleurs qu'a rappelé monsieur le rapporteur général à l'instant, cependant, cela fait des années qu'on tourne en rond sans aucune avancée sur ce sujet, donc j'espère que dans les travaux que vous annoncez, vous avez quand même à l'esprit, un moyen de contourner toutes ces difficultés, parce que sinon je crains fort que l'année prochaine on ne revienne devant cette assemblée, en nous disant que il y aura des livraisons à partir d'entrepôt à l'étranger, il y aura des contournements c'est pas faire la différence entre les biens livrés dans le cas du E-commerce à partir des entrepôts et les biens qui vont dans le commerce traditionnel, et donc je crois que Madame la Ministre, il faut que cette mobilisation générale et la créativité que vous annoncez soit vraiment respectée parce que ça commence vraiment à être très fatigant, tous les ans, d'entendre le même discours, merci. Si Monsieur Salmon pour explication de vote. Merci madame la présidente, monsieur le rapporteur, madame le la ministre, je suis aussi très satisfait, je reprendrai pratiquement mot pour mot les les propos de mon collègue Bazin effectivement moi ça fait 2 ans que je suis au Sénat 2 ans que régulièrement on redéposer le même amendement et que, hé bien, effectivement, ça ne va jamais tout à fait bien sans doute qu'il n'est pas parfaitement construit, mais il faut travailler, il faut s'y mettent à alors j'entends, j'entends vos propos donc. évitons que on se revoit dans un an, toujours dans les mêmes dispositions et que là, vraiment, on est un travail parce que quand il y a une volonté, il y a un chemin, merci. Merci, Monsieur Lemoine pour explication de vote. Merci beaucoup, madame la présidente, très clairement, il y a une volonté, elle a été exprimée par la ministre, elle s'inscrit dans la suite des Assises du commerce qui se sont tenues, il y a un an pile, et au cours desquelles justement les acteurs et on la diversité la myriade d'acteurs d'acteurs différents qui oeuvrent dans le commerce ont souhaité mieux structurer la filière, d'où le conseil national du commerce pour y conduire ce type de travaux, l'amendement telle qu'il est rédigé effectivement chers collègue on envoie un certain nombre de de limite on on pourrait se retrouver à frappé par exemple des entrepôts de Tir prestataires, est ce que on va frapper par exemple la Poste qui par ailleurs achemine un certain nombre de colis, il y a d'expédition familiale et cetera, donc je pense que il faut pour remettre de l'équité parce que ça le besoin, il est là, peut être regardé sur d'autres pistes, le collègue Bazin évoquait les livraisons ayons en tête d'ailleurs les travaux conduits dans cet hémicycle, je me souviens de Laure Darcos ce qui proposait justement pour remettre de l'équité, par exemple dans le monde du livre, hé bien qu'il y ait un prix minimum pour les livraisons, on peut s'inspirer de ce type d'initiative, je crois qu'il faut redire l'action de de la Haute Assemblée en la matière aussi ne pénalise ont pas, par exemple, le milieu rural parce que parfois, effectivement, vous pouvez être amenés à à à passer par ce type de également de prestation peut être qu'une piste, ça peut être aussi puisque Madame, la ministre a évoqué la nécessité de travailler là-dessus et donc je Live cette piste peut-être de facturer obligatoirement les retours des produits parce qu'il faut voir que 20 à 30 % des produits expédiés souvent reviennent et ça signifie que, il y a là un énorme chantier environnementale c'est dans, c'est le cas dans la ce qu'on appelle la Fast fashion, un certain nombre de de marque plutôt asiatique d'ailleurs qui utilisent beaucoup cela, donc voilà quelques pistes mais aujourd'hui, chers collègues, je pense que il faut privilégier ce travail de fond et nul doute, je vois la détermination du gouvernement que dans un an, nous n'aurons pas le débat, puisque nous aurons agit voilà madame la présidente. Monsieur le sénateur Monsieur Bocquet pour explication de vote. merci. je vais devoir me faire pardonner, je ne sais pas. Mais vous êtes vous êtes pardonnez-moi, vous avez qu'un problème hein à la présidente, madame la ministre, aussi je vous pardonne à l'avance, aussi, au cas où nous allons soutenir ce veut non je dis à mon collègue le mois des ancien ministre qui est venu à votre secours, là je le Moine, par l'exemple de la Poste. Il est mauvais, l'exemple. Vous avez parlé de Stuart c'est une filiale 100 % qui a été crée par la Poste, qui est accusé pour travail dissimulé, Monsieur Lemoine. Chers collègues. Donc, vous voyez ce qu'a dit l'autre collègue Bazin et tout à fait fondée et faut qu'on fasse attention comme on traite cette question là c'est pas donneur de leçons mais attention quoi. Et j'attire aussi votre attention chers collègues, c'est que la fameuse plateforme Stuart, qui a été créé par la Poste à 100 pour 100, est accusé aujourd'hui de travail dissimulé, mais moi je vais vous dire on va aller plus loin, aussi à la crève 20 société 20 l'E-commerce avec Stuart. Qui comme par hasard, mes chers collègues, à une activité qui est de moins d'un an. Donc pas de fiscalité. Donc, il rentre en totale concurrence avec notre économie traditionnelle notamment TPE-PME, donc vous voyez, on est sur un sujet aussi sensible que ça, donc je pense que quand on veut défendre la valeur travail, faut reconnaître le travail de ceux qui l'exercent merci. monsieur Savoldelli je mais aux voit ces deux amendements avec 2 avis défavorables qui vote pour l'amendement.

Alors cet amendement 149 de la loi des finances pour 2017 avait su se substituer aux dotations forfaitaires et dotations de péréquation des régions, une fraction du produit de la TVA, la même réforme a pourtant exclu et presse expressément la dotation de continuité territoriale du calcul, privant ainsi la collectivité de Corse de davantage de recettes dynamiques liées à la TVA sur la fraction de ses recettes, je rappellerai que la dotation de continuité territoriale est une dotation qui vient en compensation d'un transfert de compétences de l'État à la collectivité de Corse, autorité organisatrice des transports aériens et maritimes entre l'île et le continent, avec l'obligation de mettre en oeuvre les modalités permettant d'atténuer des contraintes de l'insularité aussi le présent amendement propose de revenir sur le choix peu compréhensible du gouvernement en intégrant à la dotation de continuité territoriale dans la liste des dotations remplacée par une fraction de la TVA. si, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Madame la ministre. Ce sera le même avis, madame la présidente. Vous retirer je mets aux voix.

je comprends l'intérêt bien entendu de de mon collègue, suis pas de vouloir consolider la dotation de de continuité territoriale mais je pense que vouloir la remplacer, aujourd'hui je dirais par une fraction de TVA dans le contexte économique incertain, actuellement, ce ne serait pas plus prudent et je pense que une réindexation tous les ans sur la fluctuation des des carburants sera beaucoup plus raisonnables, c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur l'amendement de mon collègue, Paris. Merci, chers collègues, je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre. Abstention : il n'est pas adopté, nous passons à l'article 11 bis à monsieur Gremillet le 1500 Oui merci madame la présidente, madame ministre monsieur le rapporteur général chers collègues. Cet amendement a pour but, tout simplement, de revenir sur les Adilia de quatre car si d'un côté, il est judicieux, effectivement, de supprimer la redevance applicable aux concessions hydroélectriques par compte revenir sur tout le travail parlementaire qui a été fait entre l'Assemblée et le Sénat, revenir sur le travail parlementaire du Sénat sur la loi sur l'hydroélectricité et d'un accord qui a été trouvé à la fois sur la loi énergie-climat de 2019 à la fois sur climat révision de 2021 absolument incroyable, donc je je propose tout simplement de revenir au texte qui a été votée sur l'hydroélectricité qui permet d'augmenter la puissance à un moment où aujourd'hui on a besoin de plus de puissance électrique dans notre pays, qui plus est décarbonnées je propose aussi de simplifier, c'est ce que nous avions décidé au niveau du sénat de simplifier, c'est ce qui avait été voté là aussi et je suis très surpris quand même qu'au travers de d'un texte sur les finances revienne sur le travail parlementaire notamment de fond sur la production d'hydroélectricité dans notre pays. Monsieur le rapporteur, votre avis. Je propose qu'on ne revienne pas sur ce travail parlementaire, c'est donc un avis favorable. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, bonjour, monsieur le sénateur Gremillet, l'article 11 bis ne prévoit pas la suppression du 3ème alinéa de l'article L. 511 Tiret 6 Tiret 1 du code de l'énergie, l'article 11 bis ne remet pas en cause. Le principe d'une décision d'acceptation en l'absence d'un délai de 6 mois renouvelable une fois, après transmission du dossier. Il renvoie à un décret en Conseil d'État pour déterminer et vous l'avez dit, les modalités d'application qui sera encore nécessaire de préciser en particulier la façon dont l'acceptation est prononcé en dehors des dispositions du silence vaut acceptation, le gouvernement envisage en effet que cette acceptation se fasse sans modification du contrat de concession, c'est-à-dire sans un avenant dans un souci de simplification de la procédure administrative telles que c'est bien prévu dans le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables à l'article 16 c'est c'est bien parce qu'il s'agit ici d'une loi de finances que l'article 11 bis ne précise pas en détail ses modalités, mais renvoie en Conseil d'État, dans ces conditions, ce sera une demande de retrait quelque part parce que votre amendement est déjà satisfait et, le cas échéant, le gouvernement aura un avis défavorable qui diverge de celui du rapporteur, mais j'espère que les explications apportées ont ont vocation quand même à vous rassurer sur le fait que le la, la procédure n'est pas bousculé, je vous remercie. Merci monsieur Rémy pour explication de vote. Oui, explications de vote, madame la présidente, madame la Ministre, j'ai bien entendu votre je voudrais remercier notre rapporteur général je maintiens cet amendement pourquoi parce que il n'est pas uniquement sur la simplification, il est aussi sur l'augmentation de de puissance, c'est-à-dire que les les lois que nous avons voté permettent effectivement au niveau des turbines au niveau des un peu le principe de ce qui a été fait sur le texte sur l'accélération des énergies renouvelables, notamment en matière d'éolien puisqu'on peut passer d'un mât de 100 mètres à 120 mètres sans qu'il y ait de nouvelles autorisations, ce que nous avons voté au Sénat sur l'hydroélectricité, c'était le même principe, c'est qu'un concessionnaire puisse augmenter la puissance hydroélectrique produite et c'est d'autant plus important aujourd'hui, Madame la Ministre, que vous savez que pour l'hiver 2022 23 les consignes qui sont données, c'est effectivement de terminer le plus possible, c'est-à-dire qu'on a donné la capacité au concessionnaire de produire un peu plus d'électricité parce qu'on en a besoin et ce que je vous propose tout simplement, c'est de continuer d'encourager les investissements d'hydroélectricité dans nos territoires énergie territorial mais aussi énergies décarbonnées. Merci, je mets donc. On voit cet amendement avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement, chers collègues, vous vouliez une explication de vote allez-y. Oui merci madame la présidente, effectivement je souscris totalement à ce que vient dire notre collègue grenier à à ce sujet, il est fort à parier, effectivement que le dispositif proposé génère un effet d'aubaine à ces problématiques en la matière sur un sujet que nous avons déjà effectivement largement débattu et j'en réfère à la proposition de loi du hein du collègue donc nous se tiendront l'amendement du collègue Rémi. on voit cet amendement avec Madame le Ministre, vous vouliez rajouter quelque chose. peu importe le résultat du vote que nous avons le même objectif, donc voilà, je vais vous le Rhodia.

Contre, abstention il était adopté article en squatter un amendement du gouvernement le 1171 Madame la Ministre. Madame la présidente, vous l'aurez remarqué c'est un amendement qui supprime de l'article 11 quater du projet de loi de finances pour 2023 les dispositions prévoyant des gages qui n'ont pas été levés lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement du gouvernement. Je mets donc aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission qui vote pour. Contre, abstention, il n'est pas adopté. Il est adopté, pardon, excusez-moi, j'étais en train de me dire que. Dimanche. Je mets aux voix donc l'article en squatter qui vote pour.

Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, cet amendement vise à ne reporter que d'un an, l'actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. C'est une demande qui est. Orthogonal à la demande de la commission des finances, qui s'est attaché à demander les deux années pour permettre, de parfaire le dispositif, dont le ministre lui-même a convenu qu'ils présentaient, de vrais imperfections après son adoption par le Parlement. Madame la Ministre. Merci madame la présidente j'aurais et même remarque que le rapporteur et même avis défavorable.

Oui merci madame la présidente, alors au PLFR du mois de juillet, j'avais déposé un amendement pour demander le report de la révision des valeurs locatives professionnel parce que cette réforme était faite en absence complète de données et donc en fait ce que je vous propose par cet amendement, c'est devenir utiliser l'outil informatique qui a été développé pour le travail sur la réforme des valeurs locatives des locaux d'habitation, de le mettre à disposition aussi des locaux professionnels, ce qui permettra d'avoir une collecte immédiate et surtout d'utiliser un même outil déjà développée et qui est prêt pour être pour rentrer en fonctionnement au 1er janvier ce qui permettra d'ailleurs ensuite de pouvoir accélérer sur le processus de de révision des valeurs locatives professionnel. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis. Alors on connaît dans cette assemblée, la pertinence, en général de des propositions et de la réflexion de notre collègue Christine Lavarde. Néanmoins, je continue de m'interroger un peu, je vais donc solliciter l'avis du gouvernement, je m'interroge notamment sur la question de la comparabilité des marchés locatifs, professionnels et particuliers, d'une part et d'autre part sur la faisabilité technique de la mesure, alors j'ai entendu Zeman d'explication de notre collègue, ce que je veux dire par là c'est qu'il faut être attentif à ne pas s'alourdir certaines obligations administratives que l'on pourrait faire supporter sur les entreprises. Merci, votre avis, Madame la Ministre, donc. Si madame la présidente, je je sais par avance que un certain nombre de sénateurs vont sourire mais. Comme votre amendement pointe un un sujet important et que c'est une proposition intéressante, je veux vous dire au nom, vous l'avez, monsieur le sénateur, mais je veux vous dire très officiellement au nom du ministre des Comptes publics Gabriel Attal qu'il va monter et il me l'a dit avant que je vous rejoigne un groupe de travail, c'est maintenant que je savais que j'aurais un accueil non mais au-delà de l'humour que je chéris, ça n'est pas une proposition en l'air, madame Lavarde, je me permets de vous transmettre l'invitation si Gabriel Attal m'en voudrait, il a prévu un groupe de travail sur ce sujet précis à compter du début d'année prochaine, et c'est un groupe de travail avec lesquels il a besoin de travailler avec les élus locaux avec les sénateurs avec les députés et c'est donc une invitation que je vous transmets compte tenu de, de l'intérêt qu'il porte à votre proposition, je vous apporte deux 3 précisions en plus peut-être pour vous éclairer, en amont de ce groupe de travail, la mesure que vous proposez ne semble pas du côté du ministère des des comptes publics nécessaires parce qu'une obligation déclarative de loyer déjà prévue par l'une des annexes de à la déclaration annuelle des résultats des professionnels et le report de 2 années de l'intégration dans les bases de résultats de l'actualisation Cenal de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels là Hervé LLP permettra si nécessaire de proposer des améliorations à ce dispositif, voici 2 explications que je vous transmets au nom du ministère des Comptes publics et je réitère la constitution d'un groupe de travail, ce sera une demande de retrait, le cas échéant, défavorable, et merci pour l'accueil que vous m'avez réservé.

comme tous les collègues qui sont ici nous siégeons avec beaucoup d'assiduité aux réunions de révision des valeurs locatives or qu'elle n'est pas ma surprise d'entendre votre réponse parce que les techniciens ont devancé le groupe de travail qui allait être mis en place par le ministre, puisque déjà dans ces réunions, on nous dit que ce serait une excellente idée que de l'étendre locaux professionnels on va un peu plus vite que vous en faites. Merci madame Lavarde, explications de vote. Ah oui, mais quand j'entends la Ministre dire qu'il existait déjà une obligation légale de déclaration, mais en fait, en quelque sorte, vous vous enfoncez comment est-ce qu'on a pu avoir dans des départements, des échantillons enfin des valeurs moyennes calculées à partir de quatre quatre donné c'est juste au-dessus du du seuil de secret fiscal franchement je comprends pas, s'il y avait déjà des outils informatiques, pourquoi est-ce que le travail n'a pas été fait en amont, donc soit c'est qu'on n'arrive pas à récolter ces informations qui sont disséminés dans des bases fiscales qui sont peut être pas directement accessibles par les outils de Bercy, là c'est un outil qui a été développé par les services de Bercy pour travailler sur les les locaux d'habitation et j'ai compris que les locaux d'habitation devraient suivre exactement la même logique de réformes que les locaux professionnels, donc là on je suis pas sûr qu'ils vont faire un groupe de travail pour indiquer aux entreprises qu'elles doivent aller rentrer une donnée, il était même possible qu'au moment elles aillent faire leur déclaration fiscale il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et que ça renvoie directement c'est juste par un pont informatique entre 2 applications de Bercy, donc ça me semble pas en tout cas du de notre ressort l'expliquer comment il faut codé pour faire ça, donc je ne sais pas ce qu'on va faire dans le groupe de travail en tout cas je ne pense pas qu'on parle de logiciels. Monsieur Richard pour explication de vote. Dis donc, je je voudrais simplement faire observer à notre collègue Christine Lavarde que il y a du travail pour ce groupe de travail puisque ce que nous avons, pardon, mais enfin beaucoup ici ont participé de près aux commissions qui viennent de conclure la révision Cenal et ont constaté qu'il y avait des hein, parce qu'il y avait de sérieux déficit d'information et que par conséquent, d'une part, nous travaillons un peu à l'aveugle et les conséquences pour les contribuables, c'est-à-dire les nouvelles fixations de valeur risquait d'être arbitraire et deuxièmement que cela interroge. Pardon, chers collègues. Les constats que nous avons fait, interroge, en tout cas c'est ma perception la pertinence même de la méthode qui a été adopté à l'initiateur au départ de la réforme que j'ai pourtant soutenu et parce que le mécanisme de sectorisation géographique comporte des biais importants et risque de créer, là aussi, une imposition non conforme aux principes de prise en compte des des des facultés contributives je suis favorable à la au déclenchement du report de 2 ans de l'application de la révision, mais je pense que il ne sera pas simplement utile ce délai à perfectionner la collecte de données statistiques manifestement insuffisant insuffisant de l'heure actuelle, mais probablement à revoir aussi la méthode de concentration des données et de fixation des valeurs. Merci, monsieur le rapporteur. je pense qu'on peut travailler ensemble. Donc de partir sur le groupe de travail me va bien, l'Avantage, même en étant éloigné Christine Lavarde ne confirme, mais j'entends ce que vient dire le sénateur Richard on peut quand même convenir. je dirais d'un d'un recul sur un texte qui avait été adopté mais dont on voit avec la révision sexe anal dont on voit en fait les difficultés pour tout vous dire madame la Ministre, moi j'ai fait aussi partie, comme on a eu la faculté puisqu'on fait partie de ces commissions départementales de révision des valeurs locatives des locaux professionnels et j'étais. Toujours assez admiratif de l'optimisme des services qui ont conduit les démarches puisqu'en fait on s'aperçoit selon les départements, et d'ailleurs, en théorie, parfois ça fonctionne bien, c'était plutôt les éléments dont on avait, nous, eu à connaître et je le dis, on s'était plutôt entendue, il a juste me semble-t-il, toujours une difficulté, c'est que, comme c'est très théorique que c'est fait globalement à marche forcée, donc on est quelques-uns, on écoute les propositions des services de l'État et on regarde les cohérence générale, par contre, on n'a pas du tout de matérialité dans la transformation pour voir les coûts et surtout ce qui me paraît aussi préjudiciable, c'est que dans la démarche, on passe par des commissions ensuite de révision des valeurs locatives qui se qui doivent se tenir en plein été, parce que le calendrier est très resserré pour les phases de validation, c'est-à-dire que, en gros, personne n'a le temps de se pencher vraiment sur la question, à part les quelques uns qui sont réunis autour des services départementaux des des voilà donc je pense, pour aller un peu plus loin que le groupe de travail est un début, vous l'avez proposé en entrée ou la proposant sortie donc je me rangerai à cette proposition, et donc un avis de retrait au bénéfice du groupe de travail. Madame Lavarde vous retirer alors je mets aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour.

donc le vingt-neuf, président de l'Haye. Oui, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors moi je suis madame la ministre. Candidat pour être faire partie du groupe de travail qui devrait avoir du travail, si j'ai bien compris donc ça m'intéresse aussi, effectivement, cette révision des valeurs locatives sur les locaux professionnels et là mon amendement concerne et les locaux d'habitation dont les valeurs locatives remonte aux années 70, dont on connaît tous un peu les les écarts qu'on peut constater chez un et chez les autres aujourd'hui et dont la révision générale était prévue pour 2000 vingt-six serait repoussée à 2028 en tout cas, on sent bien que personne n'a le courage, en fait, de se lancer dans une révision générale qui risque de bousculer beaucoup de choses, donc, à défaut de cette révision générale, j'ai une proposition que j'ai déjà formulées, qui avait déjà été adopté ici au Sénat, qui était de réévaluer en fait les valeurs locatives au fur à mesure des mutations, que ce soit effectivement des des ou des successions, que l'on puisse progressivement faire cela, alors ça prendra du temps, c'est vrai que on aura peut-être quelque chose à jour dans 40 ans, mais au moins, au moins on aura entamé le processus et, progressivement, ça peut se faire sans trop de douleur et sans avoir besoin d'un courage extraordinaire pour le faire. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis. Ce sera sur un sujet qui est, effectivement, on a parlé des valeurs locatives des locaux professionnels, les valeurs locatives concernant effectivement les habitations c'est aujourd'hui. un constat, c'est qu'il y a des inégalités criardes et ce que propose le sénateur de Haye qui a l'habitude d'avoir toujours des positions 13 apaisé modéré tout en équilibre, mais là, en tous les cas bien tranchée sur la proposition de conduire cette réflexion, moi j'ai envie de dire madame la ministre, un avis de sagesse pour quand même nous inviter à travailler ensemble à avancer sur ce sujet parce qu'à force de tourner autour du pot et de ne pas prendre de décision finalement, y compris les collectivités territoriales se retrouve en décalage et parfois en difficulté à gérer des de véritables inégalité les valeurs locatives mérite en tous les cas, notre attention, alors je pense que la difficulté, là, c'est de faire à chaque mutation mais c'est une difficulté en même temps c'est ça peut être une opportunité. Merci madame la ministre. où on peut élargir celui d'avant, c'est une invitation. Non, la révision au fil de l'eau que vous proposez, monsieur le sénateur, elle consisterait donc à actualiser la valeur locative lors de chaque changement de propriétaire, voire de chaque changement d'occupant elle ferait donc coexistent et en réalité de catégories différentes de base, elle présenterait un risque constitutionnel que je me dois de mentionner de rupture d'égalité entre les contribuables, j'ajoute que la complexité de la mise en oeuvre d'une telle procédure pourrait nuire à la lisibilité à l'acceptabilité de cette réforme est en définissant pas précisément comment pourrait être calculé la valeur locative à mettre à jour avant la mutation et donc en réalité on ne définissant pas l'assiette de la taxe votre mesure pourrait être qualifié de d'incompétence négative et en cours également à ce titre, le risque d'une censure constitutionnelle dans ces conditions, je vous demanderai donc de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur de la le cas échéant, sera un avis défavorable je vous remercie. Merci, monsieur, vous aviez demandé la parole pour explications de vote. Merci madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, alors moi je, je soutiens totalement l'amendement du président Delaye parce qu'il me paraît empreint de bon sens, on voit bien avec le sujet des locaux professionnels, combien il est difficile de mener la réforme, alors imaginez la difficulté qu'il ira ensuite à réaliser celles des propriétés individuelles pour l'ensemble de nos concitoyens et donc il est temps que l'on d'avance sur le sujet et je trouve que la méthode proposée par le président de la elle est empreinte de bon sens: pourquoi, tout simplement parce que lorsqu'il y a des mutations, hé bien, on connaît la valeur de l'immeuble et donc on peut établir immédiatement une nouvelle valeur locative qui se base sur la réalité du prix des immeubles ou des maisons ou des appartements et donc je ne vois pas en quoi il y aurait un risque d'inconstitutionnalité, c'est ce que le gouvernement avance à chaque fois qu'on évoque ce sujet, mais aujourd'hui le système est profondément inégalitaire, puisque les valeurs locatives n'ont pas été révisés c'est aujourd'hui qu'il y a des inégalités justement et que le risque d'acrostiche étais devrait être mis en avant, mais je ne vois pas pourquoi à partir du moment où, où, petit à petit, on avance vers un système qui permettra d'avoir des biens des qui soient effectivement fiable, ce serait anticonstitutionnel, il y a pas de raison et et ce système a l'Avantage en plus de permettre à ce que ça ne modifie pas pour ceux qui ont payé jusqu'à présent, la taxe avec un taxe foncière, ça ne modifie rien et ce, le nouvel acquéreur qui sur la base du prix qu'il auquel il achète le le qui paye la la la nouvelle base de valeur locative donc la nouvelle taxe, en fait, donc je crois que il faut que nous soutenions ce projet que nous puissions avancer sur le sujet, sinon je pense que jamais on ne la fera, on ne fera que reporter à des jours meilleurs et jamais il y a des jours meilleurs. Monsieur Richard pour explication de vote. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, lorsque monsieur de La Haye a fait circuler son son amendement, je me suis interrogé sur l'opportunité de le cosigné et ma première réaction a été la vôtre, mes chers collègues, ça n'a que trop duré, c'est une idée intéressante que de procéder ainsi à une réévaluation de la valeur locative des locaux gré chaque mutation, on avançait, ce faisant, et c'est ce que vous voulez, en fait, je me suis rendu compte que c'était une fausse bonne idée parce qu'effectivement on allait créer ce que Madame la ministre a signalé tout à l'heure une disparité flagrante entre des propriétés de même valeur selon ce même valeur pour nous, selon qu'elle a été dont elle a été un temps donné, ou non, et donc moi je crois moi aussi je crains aussi, quoi qu'on dise qu'on dise Calvet à risque d'inconstitutionnalité, très fort, à cet égard, je le répète de propriété ayant pour nous officiellement la même valeur parce que l'une d'entre elles a été a fait l'objet d'une d'une mutation aurait une valeur locative qui pourrait être largement supérieur à une autre et je pense que on ne passera pas sans une évaluation des valeurs locatives générale des propriétés concernées à à une même époque ben je je sais bien que ça ne se fait pas mais et que c'était une façon, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure de faire avancer le schmilblick comme on dit, mais là, à mon avis, c'est une fausse bonne idée, titre personnel, je n'ai pas cosigné, je pense que je ne le voterai et L'objection à la proposition séduisante du président de la et je ne m'aventurerai pas trop sur le plan constitutionnel parce que j'ai peur que le dispositif actuelle, tels qu'ils fonctionnent des valeurs locatives n'est pas une base constitutionnelle très solide, si un contribuable grincheux est prêt à financer les frais d'avocat substantiel, aller jusqu'au Conseil constitutionnel aujourd'hui en alléguant que le dispositif n'a plus aucun lien avec les facultés contributives des contribuables, je ne suis pas sûr qu'il perdrait. Mais l'objection, elle est tout simplement dû au fait que si nous faisons une révision, elle sera fondée sur les valeurs de marché des locations actuel, c'est-à-dire que l'évaluation sera beaucoup plus élevée que les évaluations actuelles, ça peut être une multiplication, on l'a vu avec les valeurs locatives par 3 ou 4 et et nous savons bien que le jour où cette révision viendra, elle fera l'objet de toutes les mesures de freinage ou de, de, de limitation qu'on a appliqué que qui a donné lieu d'ailleurs où substantiel original de planchonnement, c'est-à-dire à la fois plancher et plafond, donc si vous avez sur 10 contribuable dans un village un contribuable qui a vu sa valeur révisée et qui elle a une valeur de base 3 fois ou 4 fois supérieure de celle de ses voisins soit vous appliquez individuellement un mécanisme de freinage ou de report de cette augmentation ou vous créez une inégalité devant l'impôt qui est assez forte, donc il me semble que votre idée, elle est valable, mais elle ne pourrait tourner que si on disait on a fixé la nouvelle valeur locative de tels le logement ou de telle maison mais on la garde en stock et on ne l'appliquera que le jour où l'ensemble des révisions auront lieu. Merci monsieur le président, la font pour explication de vote. Oui merci madame la présidente, autrement je n'ai pas tellement compris la proposition du groupe de travail tout à l'heure de la ministre, autant là je trouve qu'il y avait matière à proposer un groupe de travail, quelle est la question posée par le la proposition du président de la c'est pas tellement le le problème de la constitutionnalité, c'est pas ça, c'est de dire : faisons attention à cette taxe foncière afin que, on ne se retrouve pas dans la même situation dans quelques mois, que celle que nous avons connu avec la taxe d'habitation où à force de la dénoncer pendant des années en disant ce n'est pas un outil efficace et équitable, on se retrouve devant une décision qui nous est imposée parce qu'on n'a pas su par nous-mêmes la réformer, alors c'est ça que propose le le le président de la c'est que nous travaillons à cette question de la taxe foncière qui est désormais le seul impôt dont bénéficient les collectivités locales quasiment et et qui est un un un un impôt inéquitable, on le sait tous, il est économiquement contestable et il est par rapport à nos contribuables inéquitable, je me faisais la remarque en écoutant la proposition du président de lait, quelle serait la pertinence de la TVA, si elle était assise non pas sur la valeur réelle des biens, mais sur la valeur administrative évalué en 1970 quelle serait la valeur d'une TVA acquittée sur sur la baguette, si on l'évaluer, non pas au prix de la baguette aujourd'hui mais ce ce, celle de la baguette en 1970 c'est ça, la taxe foncière, aujourd'hui c'est pour ça que la proposition du du, du, du président de la certes, effectivement il faut l'affiner, il faut là mais ça le mérite de de lancer cette question il ce débat sur l'évolution de la taxe foncière, parce que si on ne le fait pas par nous même, un jour, ça ne sera imposée par d'autres et donc moi je voterai l'amendement du président de l'année.

et ça répond à notre collègue Richard n'est pas satisfaisante du tout parce que, en fonction de la date de construction des des bâtiments, même dans une même rue, on a des différences considérables de valeur locative, donc ça existe déjà le le le problème soulevé et déjà existants, donc autant se mettre en route, alors après, peut-être qu'il faut adapter certaines dispositions peut-être que et et c'est là où je rejoins président là font aussi, il y a que des présidents ici, mais le président là font qui proposait un groupe de travail mais c'est vrai qu'on peut avancer, on peut avancer sur ce sujet de façon à ce qu'on ait une réforme progressive qui soit plus indolore et qui demande moins de courage à nos gouvernants pour pour la mettre en oeuvre. Merci, je mets donc aux voix cet amendement avec un avis de sagesse de la commission défavorable du gouvernement qui vote pour.

vote contre. Qui s'abstient-il être adopté chers collègues. Juste de vous préciser que nous suspendrons nos travaux à 13 heures article 11 hommes Thiès trois amendements identiques de suppression madame Lavarde le l'amendement numéro 4. Oui, merci, je me souviens que à mon arrivée dans cet hémicycle en 2017, le 1er projet de loi de finances que j'ai eu à étudier porter sur la suppression de la taxe d'habitation au principe au prétexte que cet impôt était injuste, il y a quelques instants, le ministre Richard vient de nous indiquer qu'effectivement les aujourd'hui les valeurs locatives pourrait souffrir d'un d'inconstitutionnalité, si jamais elles étaient attaqués devant le Conseil constitutionnel alors est-ce à dire Madame la Ministre, que par ce report de la réforme, vous nous annoncer un scoop, à savoir que vous allez supprimer la taxe foncière, au prétexte que cet impôt est aussi injuste pour les mêmes raisons que la taxe d'habitation parce que, même cause, mêmes effets, parce que sinon, en fait, je ne comprends pas, aujourd'hui, on vous a demandé au PLFR de juillet, le report de la révision des valeurs locatives professionnel pour une absence de données et pour une méthode définie par la DGFIP, qui était difficilement applicable ou, en tout cas, qui donnait des résultats qui n'était pas cohérent avec ce qu'on a observé sur le terrain là pour la révision des valeurs, des locaux d'habitation, on a 3 ans pour le faire entre 2023 et 2026 vous avez un outil de collecte de données qui a été évoqué précédemment, qui va entrer en vigueur au 1er janvier donc, expliquez-moi ce qui s'opposent au fait que nous commencions à travailler dès 2023 à la réforme, pourquoi est-ce qu'il a besoin de reporter comme je pense qu'il y en a aucune des raisons, c'est pour ça que je demande la suppression de l'article onze. monsieur le rapporteur, l'amendement 135. C'était, c'est exactement pour les mêmes raisons que la commission a porté un amendement identique. Monsieur Savoldelli, le 800 Remarquable de l'administration, donc c'est bien aussi de le dire aussi l'hémicycle du point de vue des services de de l'État, mais là, voilà, il faut des explications, je trouve que ce qu'a dit Christine Lavarde et le rapporteur général et dans le même état d'esprit de notre amendement, il nous faut des explications pourquoi il y a un tel report, ça doit être justifié et argumenté, voilà, il y a la question des locaux professionnels, pourquoi rien sur les locaux d'habitation. Voilà, donc, oui, si on a les explications, on pourrait éventuellement revenir sur votre position, mais sinon il faut supprimer cet article bien évidemment. Merci madame la Ministre pour avis. Merci madame la présidente. Soit je vous lis la vie soit je vous donne directement l'atterrissage hein, sans mentionner, le groupe de travail, je vous dirais jusqu'en cohérence avec le report de l'actualisation des valeurs locatives pour les professionnels, il semble logique de décaler, celle des locaux d'habitation qui est confronté, et vous le savez, à des problématiques très similaires et c'est aussi l'occasion de réaffirmer la volonté du gouvernement de conduire la révision des locaux d'habitation, comme la loi le prévoit, position qui a d'ailleurs été réaffirmé auprès de l'ensemble des associations d'élus, l'AMF bien sûr l'ADF franche urbaine et donc ce sera une demande de retrait ou un avis défavorable sur cet amendement qui dont l'objet sera aussi discutée oh, ça, je ne dirais j'ose même plus dire le mot, vous ferez la conclusion vous-même, je vous remercie. Monsieur Laménie pour explication de vote. Oui, mais merci madame la présidente, madame le Ministre, chers collègues, très rapidement concernant ces trois amendements que je soutiendrai un un amendement de suppression de l'article 11 oct séché un petit peu référence parce que les valeurs locatives, c'est très très compliqué ce c'est régulièrement rappelé bon au niveau des du calcul des bases d'imposition je ferai référence à la composition des commissions départementales des valeurs locatives et précédemment, on a longuement parlé aussi pour les valeurs locatives des locaux ça vous pour la composition des de ces commissions départementales des valeurs locatives avec 10 représentants des collectivités territoriales, des représentants du même ordre en nombre une dizaine des représentants des contribuables et de représentants de l'administration fiscale pour avoir participé comme beaucoup de collègues à la aux réunions de ces commissions départementales valeurs locatives, en particulier pour les locaux professionnels, il se trouve que se poser souvent un problème de quorum, même s'il y a des suppléants pour pour les autres représentants et les et souvent je, je, j'étais seul comme parlementaire, dans les Ardennes et il se trouve que

membres mais nous n'entrons pas en prise en compte dans le quorum donc ceux qui peuvent poser problème ça reporter aussi les les réunions, donc voilà moi c'était aussi mon interrogation et je soutiendrai néanmoins ces amendements. Merci monsieur Karoutchi Monsieur Président Karoutchi pour explications de vote. madame la présidente, pardon, Madame la Ministre, on parle souvent de la nécessité de moderniser, bon très bien, et vous parlez souvent au gouvernement de d'écouter le terrain d'écouter les remontées de terrain alors sur les valeurs locatives sur les locaux professionnels, tout le monde a acté le rapporteur général en premier qu'effectivement il y avait beaucoup de difficultés techniques, mais sincèrement, j'aimerais que plutôt que de nous dire : ah bah c'est compliqué ou ou plutôt que nous proposer un énième groupe de travail, vous nous disiez quelles sont réellement les difficultés absolu sur les valeurs locatives sur les locaux d'habitation parce que ce qui nous remonte des maires des des communes et tout, c'est que c'est faisable, franchement, ça fait des années qu'on parle de cette révision, si quelqu'un s', mais pas un jour, ça sera jamais parce que très sincèrement nous proposer un groupe de travail en 2023 c'est pas sérieux puisque vous voulez être proche des remontées de terrain, on a accepté le report sur les valeurs locatives des locaux professionnels accepter qu'on avance sur les les valeurs locatives des locaux d'habitation, je crois que ce serait bien et pour le gouvernement et pour nos collectivités. Merci monsieur Savoldelli pour explication de vote. En a merci madame la présidente, madame la miss mes, mes chers collègues. Pourquoi on on insiste. Et de manière collégiale, ici, c'est que ça fait partie des dispositions. De report. Que vous avez décidée sans débat. Via le 49 3 et et on a cette démarche qu'on a depuis le début de de l'examen de la loi de finances par le par le Sénat. Donc je vous, je vous dis, Madame la Ministre, là il y a un double problème, c'est que il y a le 49 3 2022 mais vous appliquez un autre 49 3 et là, moi, ça me pose énormément de problèmes pour le groupe communiste. C'est sur la loi de finances de 2020, parce que la décision de la révision des valeurs locatives d'habitation comme de professionnels était une décision de la loi de finances de 2020, donc ça fait un double 49 3 1 49 32 1022, à l'Assemblée et dans nos débats ici au Sénat et ça fait aussi un 49 3 sur les décisions qu'on avait pris à la loi de finances de 2020. Donc c'est quand même un vrai problème de contrat de confiance entre l'État et le travail parlementaire. Oui, madame la ministre, il y a, il y a quand même une différence entre la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et c'est des locaux d'habitation, les locaux professionnels, c'est une actualisation sexe anal qui est prévu par les textes. Les valeurs locatives des locaux d'habitation, c'est une raie vie Zion et de prendre ou de vouloir prendre du temps, 3 ans pour tenter de trouver un chemin et surtout d'avancer beaucoup plus concrètement. On a du temps devant nous. Je pense qu'on peut convenir d'une méthode, ce qui offre ou offriraient pour tout le monde pour l'État pour que l'activité pour nos concitoyens, au moins de la lisibilité et surtout de la visibilité pour aboutir à une solution qui soit plus juste, c'est la raison pour laquelle on pense même si c'est, on sait très bien que ça, il y aura des embûches, y aura des obstacles mais c'est pas en voulant les contourner ou en faisant un refus de saut d'obstacles qu'on avancera pour résoudre les différences qui ne se justifie plus aujourd'hui. Merci. Madame Lavarde. Oui, en fait, le groupe de travail, on l'a déjà puisqu'on a 3 ans pour préparer la réforme 2023 2026 donc, on a même le temps en 2023, si vous le souhaitez, de commencer notre réflexion par un groupe de travail pendant que les particuliers commencent à renseigner leur valeur locative dans le fameux outils dont on a discuté tout à l'heure et sur la base de ces informations, parce que je veux bien qu'on réfléchisse dans le vide, mais on a quand même besoin de données chiffrées pour savoir où on va pour essayer de voir ce qui va se passer si on applique la même méthode que pour les locaux professionnels ou locaux d'habitation, si on commence pas un tant soit peu à rien faire, les outils dont on va avoir besoin pour réfléchir, on n'y arrivera jamais, puis là vous reporter en 2025, vous pensez vraiment qu'on va s'attaquer à la révision des valeurs locatives à un an des élections municipales, j'en suis pas certaine, donc il est urgent de commencer à réfléchir. Merci, je mets donc aux voix ces amendements avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui vote pour. Oui, dont l'amendement de commission Titan qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient ils sentent adopté, il fait tomber le 1256 et supprime donc cet article à l'amendement 628 monsieur

pour jusqu'à maintenant, les équipements nécessaires à la méthanisation bénéficiaient de même type d'exonération, il s'agit de production différentes de production agricole, il paraît donc légitime de revenir sur cette exonération, ce qui générait des ressources aussi pour les communes rurales qui accueille ce type d'installation qui génère des charges en particulier des charges de voirie. Madame la Ministre. J'aurais le même avis, madame la présidente. Je mets donc aux voix ces deux amendements avec 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous passons 2 amendements identiques, le 498 Monsieur kaput. Merci madame la présidente, il s'agit d'un amendement qui vise à donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d'appliquer au méthaniseur dit non-agricoles, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévue pour pour la meunier totalisation agricole il s'agit donc d'apporter un soutien fort au développement de l'ensemble de la filière méthanisation, pourvu que les collectivités prennent l'initiative de se saisir de ce levier fiscal qui est placé à leur disposition. Merci, monsieur le rapporteur, ah mais attendez, non, il y a un autre amendement et Dati identique, monsieur le Président, Ruquier parfait, donc Monsieur le le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements identiques : retrait, Madame la Ministre. Merci madame la présidente, exonérés de type d'établissement que les établissements agricoles irait en réalité bien au-delà de l'incitation actuel en faveur des exploitants agricoles pour métallisé leurs déchets dans une logique de proximité et de lutte contre la pollution agricole compte tenu du Champ très large de votre proposition, votre mesure conduirait en réalité à accorder une subvention injustifiée à des entreprises industrielles, a priori, rentables et bénéficierait notamment à certains très grands acteurs du secteur, qui en réalité n'ont pas besoin d'un soutien public pour mener à bien leur activité par ailleurs ces installations, elles sont dans la très grande majorité des cas, des établissements industriels au sens foncier et elle bénéficie de l'allégement de fiscalité sur les impôts de production instauré pour 2021 par l'article 29 du PLF avec une division par 2 de leurs bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, cette mesure c'est un un soutien important au secteur industriel, il n'est pas envisagé, à cette heure d'aller au-delà et dans ces conditions, sur cette sur ces deux amendements, ce sera comme le rapporteur, une demande de retrait sinon un avis défavorable je vous remercie. Merci monsieur Camus. Oui, je précise que c'était seulement si la collectivité le souhaitait mais je compte tenu des compte tenu des Très bien, je vous remercie, cher collègue, nous passons à l'amendement 499 monsieur kaput. Alors il s'agit d'un amendement qui a pour objet de donner aux collectivités territoriales toujours celles qui le souhaitent la possibilité d'exonérer certains réseaux de chaleur de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, ces réseaux de chaleur concernés sont soumis à un double critère d'une part livré moins 10 GWh et d'autre part être alimenté à plus de 70 % par des énergies renouvelables et de récupération, je précise que, dans son rapport de septembre 2021 sur le chauffage urbain, la Cour des comptes, constatait que le mode de chauffage, réseau de chaleur était une contribution efficace à la transition énergétique qui reste insuffisamment exploité. Merci le ML n'est pas défendu le 1310 présidents Ruquier. Parfait, monsieur le rapporteur. on avait 3 identique, puis à 1088 je ne voudrais pas vous priver de parole monsieur ça me je faire pardon. Oui, pour compléter c'est si si l'installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste, ils sont en revanche actuellement confrontés un équilibre économique fragile, une application des impositions locales aux réseaux de chaleur aurait des conséquences, des conséquences financières très compliqué sur les charges du service et, in fine, et sur les tarifs facturés aux abonnés par ailleurs l'assiette et les taux de ces impositions sont variables d'un site à l'autre, ce qui, par rapport au chiffre d'affaires dans le service public pourrait représenter un poids de 2 à 10 % en fonction des réseaux il faut le préciser, ne vise pas exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces imposition mais à circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions aurait un impact trop important sur leur compte et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Merci donc monsieur le rapporteur, notre avis sur ces 3 hommes.

aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'installations qui sont extrêmement vertueuse qui ont trouvé leur équilibre, elles sont en régie sont en délégation de service public, elles sont concédées, enfin peu importe mais dans au moins dans ces cas-là dans le modèle de l'entreprise dans le l'équilibre financier, évidemment les charges liées à la fiscalité du site sont intégrés et comme progressivement. L'ensemble des réseaux de chaleur. Notamment les plus vertueux, mais ils vont tous devenir l'objectif, c'est qu'ils répondent aux orientations de lutte contre le réchauffement climatique et de réduction de l'impact de la pollution dans l'air. Je ne comprends pas et je ne vois pas la logique de vouloir. Proposez certes d'offrir la faculté d'exonérer des enfin ces dispositifs au détriment des recettes des collectivités locales en fait il faut parce que sinon ça veut dire qu'à terme, le jour où la société et pourquoi le faire plus pour ces dispositifs, mettons que pour une entreprise publique, dans un cas, une entreprise privée, une entreprise associative qui s'inscrit dans une même démarche avec des locaux extrêmement vertueux de bâtiments passifs, on pourrait dire : bah, écoutez, non pas de consommation énergétique en en excellente environnement, respect de la biodiversité, sur le site on exonère mais alors va chercher ou les recettes, voilà, c'est ce qui m'invite à 4 demande de retraite. Merci madame la Ministre même avis. J'aurais oui, madame la présidente, le même avis que monsieur le rapporteur, je voudrais juste donner de chiffre pour éclairer la représentation nationale, le budget du fonds chaleur c'est en 13 ans plus de 3 milliards d'euros d'investissement ce budget du fonds chaleur, il a d'ailleurs récemment été augmentée et portée à 370 millions d'euros sur la période 2009 2021, ce fonds a soutenu plus de 6500 opération le rapporteur l'a rappelé son action s'inscrit dans les objectifs structurels de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sont eux-mêmes fixé à plus de 25 % de chaleur renouvelable en vingt-trois et entre 40 et 60 en 2028 par rapport à 2017 pour les autres raisons et notamment le le point d'incohérences soulevées par le rapporteur, le gouvernement aura le même avis que le rapporteur demande de retrait sinon un avis défavorable sur ces amendements, je vous remercie, madame la présidente. Je vous en prie.

Nous votons donc avec 2 avis défavorables, amendement 1088 qui vote pour. Contre, abstention, il n'est pas, z'adopté. 3 amendements identiques, le 516 Monsieur

on est donc dans une problématique totalement différente, il permet ainsi d'établir une équité de traitement avec les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche exonérés de plein droit du paiement de la taxe foncière, au titre de l'article 1382 du CGI l'exonération proposée ici s'établit à l'initiative des collectifs invité territoriale. Pour l'enseignement supérieur non lucratif et la recherche, ces établissements soutiennent en effet l'économie locale, l'attractivité territoire et le dynamisme des bassins d'emploi. Merci madame Vermeillet, amendement 532 identique merci madame la présidente. Très bien défendue par Emmanuel Capus mais j'insiste sur le fait que c'est une possibilité, et que cet amendement est à l'initiative des collectivités territoriales, c'est une liberté qu'on leur laisse dans l'esprit du débat qu'on a eu hier sur la liberté d'administration merci. Merci Monsieur Piem noir amendements identiques 1000 100 58. Merci madame la présidente, pour éclairer un petit peu et pour compléter les, les, les arguments donnés par mes collègues à l'instant, je dois dire que les explique les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général d'abord contribue à la diversification des formations sur les territoires 1er point et ensuite elle bénéficie d'un Label dans la Belle national qui est décrété qui est donné par l'État, l'intérêt général, ça leur donne des des obligations, notamment en terme d'accueil d'étudiants boursiers notamment d'accueil aussi d'étudiants en situation de handicap, ils sont souvent pointées pour pour ces ces, ces, ces bonnes conditions d'accueil. Mais.

c'est moins de 6 % de ce que coûte un étudiant en enseignement public et c'est bien là le l'objet de cet amendement, c'est de, non pas de compenser cet écart que moi même je je je plaide hein pour pour compenser une partie de cet écart à chaque rapport pour avis que je que je que je commets en commission culture, éducation, communication, mais en tout cas là de donner la possibilité de renforcer le lien territorial entre les collectivités territoriales et les écoles qu'elles accueillent sur leur territoire, via un processus qui est facultatif puisque, comme l'ont dit, nos collègues, c'est une possibilité qui est offerte aux collectivités territoriales d'exonérer sur la taxe foncière et ça sécurise le soutien de ces collectivités territoriales à leurs écoles puisque ça évite d'avoir chaque année à examiner une une dotation qui peut faire l'objet de on le sait bien, de, de, de débats parfois un peu long et et un peu superfétatoire, donc ça ça ça ça donne de la perspective aussi à cet établissement supérieur d'intérêt général, rappelons-le. Merci, votre avis, monsieur le rapporteur. Triple avis de sagesse. Madame la Ministre. Merci madame la présidente, sur ces amendements, la différence de traitement entre établissements d'enseignement supérieur, public et privé, justifiés par le caractère non productif de revenus des premiers dans la mesure où les établissements privés, y compris ceux d'ailleurs à but non lucratif sont productifs de revenus, il se trouve dans une situation différente et donc logiquement soumis à la taxe : la taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt réel du otite de la détention des biens immobiliers, indépendamment de l'affectation de la qualité du propriétaire et tout régime dérogatoire doit être strictement justifier l'exonération des établissements d'enseignement privé entraînerait des demandes similaires de la part d'autres organisme priverait qui, sous une forme ou une autre, quelque forme que ce soit participer à l'exécution des services publics, les collectivités territoriales peuvent tenir compte des impôts acquittés par les établissements privés d'enseignement supérieur via les subventions si elle souhaite soutenir leur développement pour toutes ces raisons, ce sera du côté du gouvernement sur l'ensemble de ces amendements, un avis défavorable je vous remercie.

d'intérêt général, je le répète, et de l'autre côté, lorsqu'on offre une possibilité aux collectivités territoriales c'est pas l'état de, de, de faire un geste pour ces écoles qu'elles accueillent sur leur territoire, c'est non également, vous l'avez dit, ça doit être justifié ça il me semble que c'est largement justifiée par la diversification des formations coffre ces ces établissements, je vous remercie. Merci, je mets donc aux voix ces trois amendements avec un avis de sagesse de la Commission défavorable du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient ils sentent adopté je vais suspendre la séance, chers collègues, elle sera reprise à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement séance suspendue bon appétit.